Monsieur le président,

Dans la discussion générale, la parole est à M. Alain Marc, auteur de la proposition de loi. Monsieur

nous avons tous, au sein de cet hémicycle, le souci d'une bonne administration locale. Si le nouveau mode de désignation des conseillers communautaires, dessiné par la réforme de 2013, est dans l'ensemble satisfaisant, certaines difficultés demeurent toutefois En effet, les conseils municipaux ont perdu la faculté de remplacer leurs délégués au sein des conseils communautaires en cours de mandat : les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci. Avant la réforme de 2013, un conseil municipal pouvait, à tout moment, remplacer les délégués qu'il avait désignés. La perte de cette possibilité peut provoquer des dysfonctionnements en cas de dissensions entre le conseil municipal et les représentants de la commune au conseil communautaire.

qu'il n'est pas membre du conseil communautaire. Ces difficultés se posent aussi bien dans les communes de moins de 1 000 habitants que dans les communes plus peuplées, puisqu'une modification de l'ordre du tableau municipal en cours de mandature n'a pas pour effet de mettre fin au mandat des conseillers communautaires en exercice. Il peut également arriver que le maire, même s'il le souhaite, ne siège pas au conseil communautaire. En effet, dans les communes de 1 000 habitants et plus, rien n'oblige le conseil municipal à élire le maire parmi les conseillers municipaux qui ont également été élus au conseil communautaire, ni même parmi ceux qui y ont été candidats ; nous en avons des exemples. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, si le maire élu au début de la mandature devient nécessairement conseiller communautaire, sauf s'il ne le souhaite pas ou s'il démissionne de ce mandat, il n'en va pas de même de ses éventuels successeurs. Afin de renforcer l'indispensable coordination entre les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est apparu nécessaire d'apporter des ajustements au mode de désignation des conseillers communautaires issu de la loi du 17 mai 2013, qui a privé les conseils municipaux de la prérogative consistant à élire les représentants de leur commune auprès de l'EPCI à fiscalité propre auquel celle-ci appartient. La proposition de loi tendant à renforcer les synergies entre les conseils municipaux et les conseils communautaires, que je suis heureux de vous présenter, a précisément pour objectif de résoudre les difficultés issues de la réforme du mode de désignation des conseillers communautaires adoptée en 2013. Pour ce qui est des communes de 1 000 habitants et plus, leur représentation au sein des conseils communautaires serait désormais assurée, d'une part, par le maire, sauf si, à la demande de celui-ci, le conseil municipal décidait de désigner un autre de ses membres d'autre part, par des conseillers communautaires élus en même temps que les conseillers municipaux au suffrage universel direct, selon le système de fléchage aujourd'hui en vigueur. Plus précisément, les électeurs d'une commune seraient appelés à élire un nombre de conseillers communautaires correspondant au nombre total de ceux qui sont impartis à la commune, mais le maire, s'il n'avait pas été élu conseiller communautaire au suffrage universel direct, prendrait la place du dernier candidat de même sexe élu conseiller communautaire sur la même liste que lui ou, le cas échéant, du seul candidat élu sur cette liste. À la demande du maire, le conseil municipal pourrait cependant désigner un autre de ses membres pour siéger au conseil communautaire à sa place. Le

ailleurs, le conseil municipal pourrait à tout moment procéder au remplacement d'un conseiller communautaire par un autre conseiller municipal du même sexe et ayant figuré sur la même liste de candidats au conseil communautaire, sous réserve qu'au moins un conseiller municipal ayant figuré sur cette liste le demande. Cette condition a pour objet de prévenir d'éventuelles pressions de la majorité sur des conseillers communautaires : la demande devrait être faite par un colistier du conseiller à remplacer. Afin de faciliter le remplacement de conseillers communautaires en cours de mandature, il est également proposé d'augmenter le nombre de candidats sur les listes. Aujourd'hui, les listes pour le conseil communautaire doivent comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'une unité, si ce nombre est inférieur à cinq, et de deux, dans le cas contraire.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires continueraient à être désignés dans l'ordre du tableau du conseil municipal, mais celui-ci pourrait à tout moment, par délibération motivée, remplacer un conseiller communautaire par un autre de ses membres pour la durée de son mandat restant à courir. Enfin, l'article 6 procédait à diverses coordinations dans le code électoral et le code général des collectivités territoriales. Je me félicite de ce que M. le rapporteur, Dany Wattebled, ait partagé les objectifs de cette proposition de loi, tout en affinant son dispositif, avec l'aide des membres de la commission et de mes chers collègues. La commission a ainsi approuvé le relèvement facultatif du nombre de candidats supplémentaires sur les listes de candidats au conseil communautaire dans les communes de 1 000 habitants et plus, prévu à l'article 5, en portant leur nombre maximal à quatre dans les communes élisant au moins cinq conseillers. Plusieurs autres modifications ont été apportées au régime électoral des conseillers communautaires, dont la suppression de l'incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l'exercice d'un emploi salarié auprès d'une commune membre. Par ailleurs, dans le même objectif de renforcement des synergies entre conseils municipaux et et communautaires, la commission a prévu l'institution d'une conférence consultative des maires dans les communautés de communes et d'agglomération, ainsi que dans les communautés urbaines, à titre obligatoire dès lors que 30 % des maires des communes membres en feraient la demande. Elle a également entendu renforcer les attributions consultatives de la conférence métropolitaine des maires de la métropole de Lyon, chère à François-Noël Buffet. Monsieur le ministre, mes chers collègues, en tant que représentants des collectivités territoriales, nous avons tous constaté que lorsque les maires démissionnaient en cours de mandat ou, hélas, décédaient, les nouveaux maires n'étaient pas forcément conseillers communautaires. Il est même arrivé

De tels faits ne devraient pas se produire ! Consolider la place des maires dans la gouvernance de l'intercommunalité apparaît primordial, puisque cet échelon a de plus en plus d'importance. Par ailleurs, je souscris pleinement aux modifications ponctuelles apportées en commission, qui viennent compléter un texte qui se veut pragmatique. C'est pourquoi je vous propose d'adopter cette proposition de loi.

la proposition de loi que nous sommes appelés à examiner aujourd'hui porte la marque de l'esprit du Sénat. C'est un texte inspiré par l'expérience de terrain, celle des élus locaux que nous sommes ou que nous avons été. C'est le fruit d'un travail d'évaluation patient et méthodique de la législation. Nous savons en effet, au Sénat, qu'il ne suffit pas de voter des textes, mais qu'il faut se soucier de leur mise en oeuvre et des effets qu'ils produisent. La fonction de contrôle et d'évaluation fait partie intégrante des missions constitutionnelles du Parlement. C'est, enfin, un texte mesuré, dont les auteurs cherchent non pas à renverser la table ou à revenir sur les réformes votées au cours des années précédentes, mais à procéder aux ajustements qui apparaissent indispensables au vu de l'expérience acquise. Chacun le sait dans cet hémicycle : le bon fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre nécessite une parfaite coordination entre les conseils municipaux et communautaires. Non seulement les communes doivent pouvoir faire entendre leur point de vue au sein des assemblées délibérantes des communautés qui les réunissent, mais il est indispensable que les maires et les conseils municipaux soient pleinement associés aux décisions prises à l'échelon intercommunal. C'est, d'une part, une condition de la légitimité de l'action communautaire, car un EPCI n'est que l'émanation de ses communes membres ; c'est à l'échelle de la commune que le lien démocratique entre les citoyens et les élus reste le plus fort. C'est, d'autre part, un gage de bonne administration locale, tant les compétences communales et intercommunales sont étroitement imbriquées. Pendant plus d'un siècle, les délégués des communes au sein des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale ont été désignés par leur conseil municipal. La situation a changé depuis la loi du 17 mai 2013 et les élections de mars 2014. Il faut désormais distinguer entre les syndicats de communes, d'un côté, qui sont administrés par un comité syndical dont les membres sont élus par les conseils municipaux, et les EPCI à fiscalité propre, et de l'autre, qui sont administrés par un conseil communautaire dont les membres sont désignés selon des modalités qui diffèrent en fonction de la population de la commune. En effet, dans les communes de 1 000 habitants ou plus, dont les conseils municipaux sont élus au scrutin de liste, les conseillers communautaires sont désormais élus au suffrage universel direct, en même temps que les conseillers municipaux et selon un système dit de fléchage qui établit une corrélation étroite entre les candidatures et les résultats aux deux élections. En revanche, dans les communes de moins de 1 000 habitants, dont les conseils municipaux sont élus au scrutin uninominal, les conseillers communautaires sont des membres du conseil municipal, désignés dans l'ordre du tableau. La réforme de 2013 est parvenue, dans l'ensemble, à un équilibre satisfaisant. Grâce aux apports du Sénat, le législateur a réussi à opérer une juste conciliation entre le principe, fixé en 2010, de l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct dans la plupart des communes et la nécessité de maintenir un lien étroit entre les conseils municipaux et communautaires. Certaines difficultés n'en demeurent pas moins. En effet, en même temps que la prérogative consistant à élire leurs délégués au conseil communautaire, les conseils municipaux ont perdu la faculté de remplacer ceux-ci en cours de mandat. Cela peut provoquer des dysfonctionnements en cas de dissensions entre le conseil municipal et les représentants de la commune au sein du conseil communautaire, par exemple à la suite d'un changement de majorité municipale. Il peut également arriver que le maire, même s'il le souhaite, ne siège pas au conseil communautaire. C'est le cas, en particulier, lorsqu'un nouveau maire est élu en cours de mandature. La proposition de loi présentée par notre collègue Alain Marc et les membres du groupe Les Indépendants-République et Territoires a pour ambition de résoudre ces difficultés. La commission des lois a souscrit aux objectifs recherchés, mais elle a estimé que certaines dispositions proposées se heurtaient à des problèmes de droit ou d'opportunité et méritaient donc d'être affinées. En ce qui concerne les communes de 1 000 habitants et plus, la proposition de loi prévoyait initialement que leur représentation au sein des conseils communautaires serait désormais assurée, d'abord, par le maire, sauf si, à la demande de celui-ci, le conseil municipal décidait de désigner un autre de ses membres ensuite, par des conseillers communautaires élus en même temps que les conseillers municipaux au suffrage universel direct, selon le système de fléchage en vigueur aujourd'hui. En outre, le conseil municipal aurait pu, à tout moment, procéder au remplacement d'un conseiller communautaire par un autre conseiller municipal du même sexe ayant figuré sur la même liste de candidats, à condition que l'un de ses colistiers le demande. Nous avons constaté que ce dispositif aboutissait à faire coexister quatre catégories de représentants des communes de 1 000 habitants et plus dans les conseils communautaires, les uns désignés ès qualités, les autres élus au suffrage universel direct ou indirect. Il ne nous a pas paru souhaitable que les conseillers communautaires d'une même commune puisent ainsi leur légitimité à des sources différentes. Par ailleurs, la commission a estimé qu'il était juridiquement impossible d'accorder au conseil municipal la faculté de mettre fin, à tout moment et pour tout motif, au mandat d'un conseiller communautaire élu au suffrage universel direct. Une telle disposition aurait mis à mal l'effectivité du droit de suffrage garanti par l'article 3 de la Constitution. C'est pourquoi la commission a jugé préférable de s'en tenir sur ce point au. En revanche, pour faciliter les remplacements en cours de mandat, elle a accepté l'allongement des listes de candidats, qui pourraient ainsi comporter entre deux et quatre candidats supplémentaires en fonction du nombre de sièges à pourvoir. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, dont les conseillers communautaires sont désignés dans l'ordre du tableau, aucun principe constitutionnel n'interdit qu'il soit mis fin par anticipation au mandat de ces conseillers. Là encore, la proposition de loi prévoyait que le conseil municipal puisse remplacer à tout moment un conseiller communautaire par un autre conseiller municipal de son choix. La commission a estimé préférable de ne pas faire coexister deux catégories de délégués de ces communes, les uns désignés dans l'ordre du tableau, les autres élus par le conseil municipal. C'est pourquoi elle a prévu qu'en cas d'élection d'un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à une nouvelle désignation des conseillers communautaires de la commune dans l'ordre du tableau. De cette façon, le nouveau maire pourra siéger au conseil communautaire s'il le souhaite, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Au-delà de la composition des conseils, la commission des lois s'est attachée à trouver d'autres moyens pour renforcer les synergies entre les communes et l'intercommunalité. Suivant une proposition faite par notre collègue Mathieu Darnaud au nom de la mission de contrôle et de suivi de la mise en oeuvre des dernières lois de réforme territoriale, la commission des lois a souhaité qu'une conférence des maires soit instituée dans l'ensemble des EPCI à fiscalité propre, dès lors que 30 % des maires en feraient la demande au cours des six mois suivant le renouvellement des conseils. Cette instance de concertation et de coordination entre les exécutifs locaux, qui n'est aujourd'hui obligatoire que dans les métropoles, a fait la preuve de son utilité. Le cas de la métropole de Lyon mérite un examen particulier.

lors d'une élection distincte des élections municipales. Les communes ne seront donc plus représentées en tant que telles au conseil métropolitain et certaines communes n'y enverront même aucun de leurs habitants. Cette situation est paradoxale, car la métropole de Lyon exerce un grand nombre de compétences en lieu et place des communes et l'exercice de ces compétences exige une coordination étroite avec celles-ci. C'est pourquoi, sur proposition de notre collègue François-Noël Buffet, la commission a prévu que seraient désormais soumis pour avis à la conférence métropolitaine des maires les actes les plus importants de la métropole et ceux qui se rapportent le plus étroitement aux compétences communales. Enfin, la commission a adopté plusieurs amendements visant à clarifier le droit électoral ou à abroger des dispositions obsolètes, parmi lesquelles l'article 54 de la loi Maptam, ainsi qu'un amendement de notre collègue Jean-Pierre Grand tendant à supprimer l'incompatibilité entre l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et celui d'un emploi salarié auprès d'une commune membre, incompatibilité qui n'a pas de justification évidente. Pour finir, je tiens à remercier Alain Marc

Monsieur le président, monsieur le vice-président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, monsieur le sénateur Alain Marc, auteur de la proposition de loi que nous examinons cet après-midi, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est la première fois que je me retrouve devant vous depuis la fin du grand débat national et de la grande tournée des maires lancée par le Président de la République. C'est le 15 janvier dernier, dans le beau département de l'Eure, a commencé. Comme vous le savez, les maires ont joué un rôle déterminant dans l'organisation du grand débat : 16 132 communes ont ouvert un cahier citoyen, et la moitié des réunions ont été organisées par des élus de la République, des élus locaux. C'est important de le rappeler,

Pendant ces trois mois, nous avons pu entendre des messages simples et clairs exprimés par plus de 5 000 élus que nous avons rencontrés. On pourrait les résumer ainsi : « Nous voulons plus de liberté, nous voulons moins de contraintes, faites-nous confiance et arrêtez de nous imposer un modèle toujours plus uniforme ! » Lors de l'annonce des conclusions du grand débat, le Président de la République a montré qu'il avait entendu les préoccupations et les propositions formulées lors de ses différents déplacements. de sa conférence de presse, il a clairement rappelé la légitimité que donne l'élection aux maires, confortant ainsi la place de la démocratie représentative. Le Président de la République s'est aussi engagé à renforcer le rôle des maires, notamment en leur donnant un statut « digne de ce nom ». Nous aurons l'occasion d'y travailler dans les jours prochains, en lien, bien sûr, avec les nombreux travaux déjà menés par le Sénat. Nous sommes impatients ! Le Président de la République a également annoncé plusieurs chantiers de réformes, dont une nouvelle étape de décentralisation qui se veut plus adaptée à chaque territoire, selon trois principes clairs responsabilité, lisibilité des compétences et cohérence du financement. Certes, il faut donner davantage d'autonomie aux élus locaux, mais il faut pour cela clarifier les compétences et les responsabilités de chacun : qui paie décide, mais qui décide assume. Le Premier ministre a annoncé, il y a quelques jours, la méthode de travail qui serait suivie. Les associations d'élus et les parlementaires vont évidemment être consultés pour travailler sur l'ensemble des mesures détaillées par le chef de l'État. D'ores et déjà, nous pouvons avancer sur certains chantiers, notamment, sur celui des irritants de la loi NOTRe, loi que j'ai combattue en tant que maire et président de conseil départemental, et, plus généralement, sur tous les irritants qui concernent le couple communes-intercommunalité ; ces irritants ont souvent été, il faut le reconnaître, Monsieur le sénateur Alain Marc, votre proposition de loi est intéressante, car elle nourrit les réflexions actuellement menées. En effet, les sujets qui concernent les communes et les EPCI devront être discutés et des dispositions proposées et adoptées au plus vite, avant les élections municipales de l'année prochaine. Les élus de 2014 font partie d'une génération convalescente qui a connu des bouleversements majeurs dans l'organisation territoriale. À cela s'ajoutait, bien sûr, la baisse des dotations de l'État. Nous ne voulons pas reproduire cela.

: l'EPCI doit être à son service, et non pas l'inverse. Le maire doit être pleinement associé à la décision et être informé de l'ensemble des décisions qui sont prises. l'EPCI : il est parfaitement légitime, car toutes les compétences n'ont pas vocation à être assumées à l'échelon de la commune. Comment imaginer que les 1 258 EPCI de France soient organisés, gouvernés et gérés de la même manière ? Ce serait absurde

Soyez patients, mesdames, messieurs les sénateurs : les choses avancent ! Faisons confiance aux élus locaux pour imaginer des solutions intelligentes à l'échelle de leur territoire. Certains veulent des EPCI très intégrés,

plusieurs dispositions de cette proposition de loi, telle qu'enrichie par les travaux de la commission, vont dans la bonne direction. Tout d'abord, je salue la permission donnée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants de siéger automatiquement- s'ils le souhaitent, bien entendu -au sein du conseil communautaire. fait des rebondissements de la vie politique locale- M. Marc l'a dit avec ses mots -, cela n'était pas toujours le cas. Nous aurions pu aller plus vite encore, ou en tout cas plus loin, en généralisant cette règle aux communes de plus de 1 000 habitants, mais cela pose un problème constitutionnel évident, comme l'a rappelé le président de la commission des lois, M. Philippe Bas, lors de l'examen du texte en commission. De même, l'accroissement du nombre de conseillers communautaires remplaçants, porté quatre, est un gage de souplesse permettant de pourvoir plus facilement aux démissions. Le Gouvernement y est donc favorable. Ensuite, la possibilité pour un conseiller communautaire d'exercer un emploi salarié dans l'une des communes membres

qui instaure une conférence des maires si 30 % de ceux-ci en font la demande dans les six mois qui suivent le renouvellement des assemblées délibérantes. C'est une excellente initiative ! Dans le cadre du grand débat national, les maires l'ont beaucoup dit ils veulent être davantage associés à la gouvernance des intercommunalités, en particulier lorsqu'elles ont grandi à la faveur de la loi NOTRe. La création d'une instance dans laquelle chaque maire est présent va dans la bonne direction ; le Gouvernement la soutient complètement.

visant à faire le bien des élus locaux ce texte ne crée des contraintes supplémentaires, ce qui irait bien évidemment à l'encontre de ce que nous devons faire. Il faut permettre cette liberté, dans la souplesse et la confiance que nous devons toujours à nos collègues sur le terrain. En revanche, mesdames, messieurs les sénateurs, deux dispositions introduites en commission constituent non pas des points de blocage à ce que le Gouvernement soit favorable à cette proposition de loi- je vous rassure tout de suite -, mais des points de vigilance qui concertation importante avec les autres parties prenantes. Il s'agit, d'une part, monsieur le sénateur Buffet, du renforcement de la conférence métropolitaine de la métropole de Lyon. Un amendement adopté en commission prévoit qu'elle se réunisse au moins deux fois par an, au lieu d'une, et qu'elle soit saisie obligatoirement pour avis dans certains cas. Indépendamment de notre appréciation sur le fond- je vous fais confiance -, il aurait sans doute été préférable de mener une concertation plus approfondie avec l'ensemble des parties prenantes, prenantes, les communes, la métropole et les parlementaires, députés comme sénateurs, quelle que soit leur tendance politique. De plus, il paraît difficile de modifier le fonctionnement de la seule métropole de Lyon

En conclusion, mesdames, messieurs les sénateurs, malgré ces quelques réserves, le Gouvernement est globalement favorable à l'esprit de cette proposition de loi, qui répond à des attentes exprimées par des élus locaux de terrain désireux de renforcer les synergies entre les conseils municipaux et les conseils communautaires.

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires. À l'origine, cette proposition de loi affichait de louables intentions, en ce qu'elle cherchait à modifier à la marge les conditions de désignation des représentants des communes au sein des conseils communautaires pour consolider le lien entre les communes le lien entre les communes et l'EPCI auquel celles-ci appartiennent. Toutefois, les modalités retenues par notre collègue étaient pour certaines discutables et pour d'autres contestables, notamment quand il s'agissait de remettre en cause le principe de l'élection des conseils communautaires au suffrage universel.

Ainsi, les articles 1 et 4, qui visaient à garantir la présence du maire d'une commune membre au sein du conseil communautaire, ont été supprimés. L'objet de ces articles nous paraissait pourtant légitime, en ce que la représentation d'une commune par son maire au sein d'une intercommunalité est essentielle pour porter la voix du territoire et peser à l'égard des autres communes membres. Pour autant, le rapporteur n'a pas voulu que coexistent, au sein du conseil communautaire des communes de 1 000 habitants et plus, des membres élus au suffrage universel direct- élus dans le cadre du fléchage

L'article 2 permettait à un conseil municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus de remplacer à tout moment un conseiller communautaire, même élu au suffrage universel direct, par un autre de ses membres de même sexe ayant figuré sur la même liste de candidats au conseil communautaire. À raison, le rapporteur a estimé qu'une telle faculté porterait une atteinte manifestement disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de suffrage garanti par l'article 3 de la Constitution. Mon groupe était lui aussi opposé à cet article, qui remettait en cause les principes du suivant de liste, de l'ordonnancement de la liste, du fléchage, donc du vote des électeurs. C'était une remise en cause grave et manifeste de la règle en vertu de laquelle un élu dont le siège devient vacant est remplacé par son suivant de liste direct. Cette règle vaut actuellement dans toutes les assemblées, sans exception. mesure aurait ainsi permis de piocher dans le vivier des conseillers municipaux, au mépris de l'ordonnancement de la liste qui aura été soumis aux électeurs. On comprenait bien la logique poursuivie par l'auteur : remplacer un conseiller communautaire qui ne serait plus qui ne serait plus dans la ligne d'un groupe, en l'occurrence le groupe majoritaire, puisque celui-ci était le seul à même d'obtenir une majorité de suffrages au sein du conseil pour mettre en oeuvre telle disposition. Il s'agissait donc de pouvoir récupérer son siège pour y placer un conseiller municipal plus en phase avec son groupe, ce que le système du suivant de liste ne peut garantir à coup sûr. La remise en cause du suivant de liste pour répondre à des contingences politiques internes au groupe majoritaire n'est pas acceptable Si un conflit survient entre la majorité du conseil municipal et les délégués communautaires et qu'il devient insurmontable, il existe une solution : la démission collective pour provoquer une nouvelle élection permettant au citoyen de trancher le différend. Au-delà des raisons politiques, on imagine très bien comment ce dispositif pourrait être utilisé pour contourner le système du suivant de liste en toute circonstance ... L'article 3, qui offrait cette même faculté aux communes de moins de 1 000 habitants, est, quant à lui, totalement réécrit. Le dispositif proposé dans le texte initial est supprimé et lui est substitué un mécanisme qui repose sur l'ordre du tableau. Ainsi, en cas de cessation par le maire de l'exercice de ses fonctions, il sera mis fin au mandat des conseillers communautaires en exercice et procédé à une nouvelle désignation en fonction de l'ordre du tableau établi à la date de l'élection du nouveau maire et des adjoints. Ce dispositif semble ainsi plus satisfaisant. On peut à ce stade s'interroger sur la pertinence du texte présenté par la commission, vidé du contenu de la proposition de loi initiale. Des dispositions additionnelles ont été ajoutées par la commission. Certes, quelques-unes peuvent sembler intéressantes. Toutefois, ni réfléchies ni approfondies, elles sont non seulement sans lien avec le texte initial, mais, en plus, sans aucune cohérence entre elles. Quelle est la pertinence du seuil de 30 % qui rend obligatoire la conférence des maires ? Quel lien ce texte avait-il à l'origine avec la métropole de Lyon ? Sur ce dernier point, mes chers collègues, laissez-moi vous faire part de mon plus grand étonnement. Pourquoi avoir fait de cette proposition de loi, sans rapport direct, un véhicule législatif pour la métropole de Lyon ? Il existe suffisamment de spécialistes de cette collectivité dans cet hémicycle pour travailler à un texte spécifique et complet sur le sujet. À mon sens, vous n'avez choisi ni le meilleur outil ni le bon moment. Nous resterons Nous resterons donc prudents sur les dispositions concernant la métropole de Lyon et attendrons de connaître le sort qui sera réservé aux amendements déposés par deux de nos collègues issus de ce territoire. Enfin, de manière plus générale, chers collègues, quel est l'intérêt de légiférer maintenant sur ces sujets particuliers ?

Beaucoup d'intercommunalités ont déjà anticipé la nécessité d'avoir des moyens significatifs pour fonctionner et pour pouvoir contractualiser ensuite avec le département et la région. Il ne faut pas oublier qu'avant la loi NOTRe la taille de certains EPCI ne permettait à ces derniers ni de mettre en place des services supplémentaires à leur population ni d'avoir les moyens d'exercer les compétences stratégiques qui étaient pourtant les leurs. Laissons ces lois produire tous leurs effets. En remettant en cause des pans entiers de ces textes ou des principes comme celui du fléchage, nous pourrions prendre le risque de déstabiliser un édifice qui a besoin de se poser et de respirer. Permettez-moi de rappeler que le principe du fléchage ne coupe pas le lien entre la commune et l'intercommunalité. Il a été instauré par le Parlement pour que les électeurs sachent qui sera susceptible de siéger au sein de l'intercommunalité, dont les décisions sont de plus en plus importantes au regard des compétences dévolues à cet échelon des collectivités territoriales. Cela n'enlève rien au pouvoir de la commune En revanche, l'absence de tout contrôle démocratique sur l'intercommunalité est problématique en raison des compétences que celle-ci exerce. Le fléchage est un compromis qui respecte l'entité communale et la transparence nécessaire à la démocratie. Si les lois Maptam et NOTRe méritent d'être clarifiées et perfectionnées, faisons-le par le biais d'un grand texte général et de fond. Alors que la majorité dénonce régulièrement, et à juste titre, l'encombrement du calendrier parlementaire, voilà une proposition de loi devenue un mini-catalogue aux mesures éparses, quand, dans le même temps, le Sénat réalise des travaux importants pour évaluer l'impact des récentes réformes territoriales, revitaliser le rôle des communes, ajuster le fonctionnement des intercommunalités, créer un véritable statut de l'élu, etc. Les propositions de loi se succèdent et, me semble-t-il, loin d'être vecteurs de simplification et de visibilité, risquent de semer la confusion, d'autant plus que, on le sait, nombre d'entre elles ont peu de chance de prospérer. Concentrons-nous sur les travaux du Sénat, afin de perfectionner les lois existantes par une approche globale et approfondie. Laissons les collectivités souffler. Laissons les élus respirer. Faisons confiance à leur capacité d'adaptation et d'innovation et à leur intelligence collective. Mon groupe a jugé qu'il n'était ni utile ni opportun de déposer nombre d'amendements sur ce texte. Nous Nous avons entendu les annonces du Président de la République concernant les collectivités, confirmées à l'instant par M. le ministre. Nous attendons donc patiemment

Éloignée pour certains, faille démocratique pour d'autres, cette dernière n'en reste pas moins un échelon devenu incontournable et incontestable pour les projets de territoire. Si le fléchage mis en place par loi de 2013 est venu ajouter un lien démocratique aux EPCI à fiscalité propre en permettant l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct, force est de constater que cela n'est pas suffisant pour légitimer l'intercommunalité. Pour corriger les effets pervers des différentes lois de réforme territoriale, comme la loi NOTRe, le Sénat agit et agit bien. Je pense notamment à la proposition de loi discutée au mois de janvier dernier visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des

Soyons objectifs : nous ne serions certainement pas ici à débattre de ce texte si le fonctionnement de l'intercommunalité était toujours harmonieux et si l'esprit de coopération qui doit présider à ce fonctionnement n'avait pas été mis à mal par des regroupements forcés, par un agrandissement inconsidéré du périmètre de nombreux EPCI à fiscalité propre et par la multiplication des transferts de compétences obligatoires à leur profit. Je tiens d'abord à saluer ce texte du groupe Les Indépendants-République et Territoires et le travail réalisé par Dany Wattebled en commission,

avait pour conséquence de porter une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du suffrage inscrit à l'article 3 de la Constitution en défaisant ce qu'avait fait le suffrage universel. Elle laissait également place à l'arbitraire du maire en cas de conflit avec des membres de sa majorité durant le mandat.

Par ailleurs, les rares fois où le maire n'est pas en tête de cette liste, il est dans la grande majorité des cas parmi les suivants dans la liste et fait partie du conseil communautaire. Nous le savons tous, la situation est tout autre pour les communes de moins de 1 000 habitants, et le maintien du régime actuel est alors davantage discutable. En effet, nous faisons face à une crise de vocation chez les maires. Eu égard aux contraintes qui pèsent sur eux, aux administrés plus exigeants, aux obligations toujours plus grandes,

Cette situation ne poserait sans doute aucun problème si nombre des leviers de décision, mais également de financement n'avaient pas été transférés à l'échelon intercommunal. Si tous les conseils municipaux, et pas seulement ceux de la ville-centre, avaient un lien plus étroit avec leur intercommunalité, nous ne débattrions pas non plus de cette nécessaire synergie entre les conseils municipaux et les conseils communautaires. Le texte de la commission des lois, en particulier l'article 3 qui permet, en cas d'élection d'un nouveau maire, une nouvelle désignation des délégués au conseil communautaire, dans l'ordre du tableau nouvellement établi, garantira à l'avenir une présence du maire s'il le souhaite au sein de l'EPCI à fiscalité propre dont sa commune est membre. Nous y sommes favorables. La disposition introduite en commission ouvrant la possibilité d'une conférence des maires sur demande d'au moins 30 % d'entre eux reçoit également notre approbation sur le principe.

et de la correction selon les thématiques, qui plus est au regard de l'urgence et de l'échéance des prochaines élections municipales. Depuis sa création, l'intercommunalité a permis de renforcer, souvent de manière pertinente, la capacité d'action territoriale. Faire ensemble ce que l'on ne peut faire seul, au service de l'efficacité de l'action publique : telle est la définition du principe de subsidiarité sur lequel se construit l'intercommunalité. L'exercice des compétences intercommunales reste donc très imbriqué avec celui des compétences communales. Aussi convient-il de veiller à favoriser une étroite association des communes et de leurs élus dans la mise en oeuvre des compétences que ces communes ont décidé, en les transférant à l'intercommunalité, de gérer ensemble et non pas de déléguer sans contrôle. Toutefois, la représentation des communes au sein des intercommunalités est un sujet fréquemment irritant qui crispe la relation entre les élus d'un même territoire, alors que l'intercommunalité doit être un espace de coopération construit sur l'intelligence territoriale et le consensus à partir d'un projet de territoire partagé. Cette situation de tension à propos de la représentation des communes s'est aggravée avec la décision du Conseil constitutionnel, qui a entravé les possibilités d'accords locaux. Ces derniers mois, nous avons constaté un désenchantement important des maires et des élus municipaux, qui ont l'impression de subir des sortes de rafales d'OPA sur les compétences communales et d'être cantonnés à un rôle de figurant. Ils perdent ainsi le sens de leur engagement. Monsieur le ministre, vous avez rappelé combien le Président de la République a découvert au cours du grand débat l'existence et l'efficience de tous ces élus locaux et des maires qui font vivre la République au quotidien. Aussi, je félicite mon collègue Alain Marc

toujours les comptables de l'efficacité de l'action publique devant les citoyens. L'intercommunalité, espace de coopération entre communes, va à l'échec.

La récente vague de démissions de maires plonge les successeurs de ceux-ci dans des situations ubuesques : n'ayant pas été fléchés dès le début pour siéger au conseil communautaire, ils ne peuvent y participer et se trouvent souvent écartés de décisions

Dans ce même esprit, mieux associer les maires grâce à une conférence des maires pour débattre des enjeux et des dossiers intercommunaux est une excellente proposition. J'émets cependant quelques doutes, mes chers collègues, sur une disposition adoptée adoptée en commission qui supprime l'incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l'exercice d'un emploi salarié dans une commune membre de l'EPCI concerné. Je crains que l'impartialité d'un tel conseiller communautaire ne soit rapidement contestée et ne fragilise la cohésion intercommunale. en tout cas par une construction collective d'un projet de territoire partagé que l'intercommunalité trouve son sens et ses meilleurs avocats en recueillant l'adhésion indispensable à son action. Cette proposition de loi s'inscrit parfaitement dans cet esprit pragmatique,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà déjà un an, nous discutions de l'élection des conseillers communautaires dans le cadre de l'espace réservé au groupe du RDSE au sein de l'agenda du Sénat. À l'époque, il était question d'abroger l'article 54 de la loi Maptam, qui prévoit l'élection au suffrage universel des conseillers métropolitains à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit au mois de Je ne saurais manquer de rappeler que ces métropoles sont avant tout des intercommunalités avec de très larges compétences en matière de développement économique, d'aménagement, d'habitat, etc.- la liste est bien longue compétences qui leur sont transférées à titre obligatoire par leurs communes membres. La principale différence avec les communautés urbaines réside dans la possibilité pour le département, la région ou l'État de transférer ou de déléguer par convention certaines de leurs compétences à la métropole. Aujourd'hui, exception faite de la métropole de Lyon, les conseils métropolitains sont composés en application des règles de droit commun fixées pour les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre. Par son vote du 18 avril 2018, le Sénat a réaffirmé son opposition à la réforme prévue par la loi Maptam, qui remettrait en cause la place de la commune comme maillon central de la démocratie locale. Comme je l'ai plaidé à l'époque, le mode d'élection actuel des conseillers métropolitains par fléchage permet de maintenir un lien de proximité entre les citoyens, les élus locaux et leurs représentants au sein de l'échelon métropolitain. Pour être efficace, la construction des métropoles doit se faire au service des communes qui les composent et non contre elles, surtout quand les métropoles sont composées de plus de 100 communes, comme c'est le cas de la métropole du Grand Paris. C'est tout le sens de l'article 10 du présent texte introduit en commission. coeur de cette proposition de loi, qui vise à apporter des réponses aux difficultés qui peuvent être rencontrées lors du remplacement, en cours de mandat, d'un conseiller communautaire, au regard des contraintes du dispositif de fléchage lors de l'élection municipale dans les communes de plus de 1 000 habitants. territoriales énonce la liste finie des structures intercommunales ayant le statut d'établissements publics de coopération intercommunale, donc dotées d'un conseil communautaire. Les établissements publics territoriaux du Grand Paris ne sont pas considérés comme tels. En conséquence, il n'est pas possible d'appliquer l'article L. 273-10 du code électoral en cas de vacance d'un poste de conseiller à la suite d'une démission ou d'un décès. territoriales, complété par le b du 1° de l'article L. 5211-6-2 du même code, prévoit uniquement les modalités d'élection du premier conseil territorial à la suite d'un renouvellement communal. Il ne dit rien des évolutions de sa composition. Si l'on relit le texte à l'origine de la codification, à savoir le IV de l'article 12 de la loi Maptam du 24 janvier 2014, on pourrait penser qu'il convient d'appliquer les alinéas suivants de l'article L. 5211-6-2 pour procéder au remplacement d'un conseiller. Deux problèmes se posent alors. D'une part, sauf à ce qu'il y ait accord politique au sein du conseil municipal, un conseiller d'opposition sortant serait remplacé par un conseiller de la majorité du seul fait de la répartition des sièges à la proportionnelle. L'équilibre du conseil communautaire ne coïnciderait alors plus avec celui qui est sorti des urnes après le scrutin municipal. D'autre part, le maintien de la parité n'est pas assuré, aucune condition n'étant imposée sur le sexe de la tête de liste pour ce renouvellement partiel.

Je dois donc me contenter de le soulever. J'espère qu'une réponse rapide sera apportée, car la démission de conseillers territoriaux est une réalité. Cet exemple illustre une nouvelle fois le mal-fonctionnement du millefeuille territorial en Île-de-France, voté contre la volonté des élus locaux.

soit réélu, et que trois jeunes sur quatre sont incapables de citer le nom de leur maire. Sans remettre en cause l'intercommunalité qui correspond en principe à un bassin de vie et qui permet d'agir à un niveau plus pertinent, le renforcement des compétences intercommunales a néanmoins fragilisé la lisibilité des responsabilités entre communes et intercommunalités. Il était donc nécessaire de consolider

et des membres du groupe Les Indépendants, qui tend à renforcer les synergies entre les conseils municipaux et les conseils communautaires. S'il faut partir du constat que la réforme du mode de désignation des conseillers communautaires, issue de la loi

Les auteurs de la proposition de loi souhaitaient pallier une certaine rigidité du système de fléchage, s'agissant des modalités de remplacement du maire ou d'un représentant de la commune au conseil communautaire en cas de dissensions graves et persistantes. Aussi, ce texte,

Elle a souhaité que, à la demande de 30 % des maires, la conférence des maires, instance de coordination présidée par le président de la communauté, devienne obligatoire.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par construction, il existe des risques de contradiction et, donc, de conflit entre les communes et les intercommunalités. Car qui dit intercommunalité dit délégation de compétences à un organisme autonome dont la vocation n'est pas-

Or c'est le cas avec les réformes imposées depuis 2010, qui vont remplacer l'intercommunalité volontaire de projet par une intercommunalité obligatoire, corsetée par la loi, et dont la vocation finale est de remplacer les communes. Voilà le cap des intercommunalités dont la composition des conseils résulte à 90 % de l'application de règles imposées et non de négociations, posant ainsi la question de la représentation des petites communes, voire parfois des communes Les intercommunalités ne sont plus des coopératives de communes constituées pour exercer à plusieurs les quelques compétences que les communes ne pouvaient exercer seules, mais les substituts de communes vidées progressivement de leurs compétences essentielles.

communautés sont pourtant censées représenter les intérêts, et à une probable multiplication de propositions de loi pour tenter de régler les difficultés nées de cet état de fait. Tel est d'ailleurs l'objet du texte soumis à notre examen, qui retient quelques propositions que je qualifierai de « lubrifiantes La première consiste à rétablir, pour les communes de 1 000 habitants et plus, la désignation par les électeurs des représentants des communes au conseil communautaire, ce qui n'a rien à voir avec l'élection de représentants des électeurs, tout en fluidifiant le système par l'allongement de la liste des candidats au conseil communautaire. deuxième mesure vise à abroger l'article 54 de la loi Maptam qui prévoyait que le renouvellement général des conseils des métropoles, lors des prochaines échéances, s'effectuerait au suffrage universel direct, ce qui transformait les métropoles en collectivités territoriales. Par ailleurs, le texte officialise, quand elles existaient déjà, ou crée, quand ce n'était pas le cas, des conférences communautaires des maires. Si je vous dérange, dites-le S'agissant des agglomérations, la proposition de loi donne des pouvoirs supplémentaires à la conférence métropolitaine prévue par la loi. Cette conférence, qui se réunira désormais au moins deux fois dans l'année, sera obligatoirement saisie pour avis de tout

projets de délégation ou de transfert d'une compétence à une personne publique autre qu'une commune, ce qui est au moins aussi important. Je veux dire mon regret que l'élan purificateur de la commission ne soit pas allé jusqu'au remplacement de l'actuel mode de désignation des délégués des communes de moins de 1 000 habitants selon l'ordre du tableau,

important de rappeler une nouvelle fois combien nous sommes attachés aux territoires, à leur cohésion et au bon fonctionnement de leurs instances politiques, et combien il est essentiel pour notre pays- cela n'est pas

Nous nous félicitions donc de contribuer à améliorer leur représentation dans le cadre de cette proposition de loi. Être sénateur, c'est être et rester au contact des collectivités territoriales. Cela permet de détecter, ce qu'a fait Alain Marc avec talent, les difficultés qui peuvent survenir entre un conseil municipal et un conseil communautaire.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec un peu moins de 36 000 communes, la France fait figure d'exception en Europe. Nous constatons chaque jour la force de l'identité communale et l'importance de la commune en tant que cellule de base de la démocratie. où les hommes politiques sont mal vus, seul le maire fait encore figure d'exception et échappe aux jugements péremptoires. Pour les Français, la démocratie et la proximité vont de pair. Pourtant, les réformes territoriales successives ont renforcé le degré d'intégration des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, en leur octroyant de nouvelles compétences. L'attribution de ces nouvelles compétences obligatoires s'est souvent faite au détriment des communes et des départements, allant parfois à contre-courant de la demande de proximité tant réclamée par nos concitoyens. C'est pourquoi il est essentiel de veiller aux synergies entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, pour ne pas démunir davantage les maires. Ces synergies passent nécessairement par une meilleure implication des communes au sein des EPCI. Le maire doit avoir les moyens de répondre aux attentes légitimes de ses administrés. Sa présence au sein du conseil communautaire se révèle par conséquent bien souvent indispensable, afin d'éviter toute dissension entre ce qu'il souhaite pour sa commune et les projets de son intercommunalité. En effet, un maire empêché de siéger au conseil communautaire aura moins de prise sur les affaires qui concernent sa commune. Mes chers collègues, je souhaite également revenir sur un projet de réforme régulièrement évoqué : celui de faire des EPCI, notamment des métropoles, des collectivités territoriales à part entière, dont les conseillers communautaires seraient directement élus lors d'une élection spécialement prévue à cet effet. Ce serait alors la fin de la coopération intercommunale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les conseils communautaires sont à l'heure actuelle des outils de coopération et d'investissement au service de l'intercommunalité. Ils ne doivent pas devenir devenir des outils au service d'ambitions politiciennes : la coopération ferait alors place aux égoïsmes et aux intérêts partisans. Si un tel projet voyait le jour, loin de rapprocher nos concitoyens de la politique, il les en éloignerait davantage. Le maire deviendrait alors impuissant, et pour les investissements nécessaires au développement de sa commune, il se trouverait entre les mains d'un conseil communautaire sur lequel il n'aurait aucune prise. Pis encore, les conseils communautaires seraient alors en proie aux querelles politiciennes, là où seul l'intérêt général devrait prévaloir. Nous le savons, les trottoirs d'une commune ne sont ni de droite ni de gauche. Quand ils sont abîmés, il faut nécessairement les refaire, peu importe la couleur politique du maire. Aujourd'hui, la réfection de la voirie est un objet de négociation entre le maire et le conseil communautaire. Si les EPCI devenaient des collectivités territoriales à part entière, on pourrait légitimement craindre que le maire n'ait plus voix au chapitre en ce qui concerne les intérêts de sa commune. Vous l'avez compris, l'essence même d'un EPCI est d'être un outil d'investissement au service d'une intercommunalité et des communes qui la composent. Ces communes se rassemblent pour partager un destin commun dans l'intérêt de leur territoire. La proposition de loi tendant à renforcer les synergies entre les conseils municipaux et les conseils communautaires va dans ce sens. Elle accorde une large place au maire et préserve l'intérêt communal. Elle comporte des solutions raisonnables pour remplacer un maire en cas de démission, ou pour remédier aux dissensions apparues au sein d'une équipe. Si le fléchage des candidats a permis de donner aux conseils communautaires une meilleure visibilité démocratique et de tendre vers davantage de parité,

Dans la continuité du rapport sur les conditions d'exercice des mandats locaux, qui avait suscité plus de 17 500 contributions des élus dans les territoires, nous avions souhaité répondre au sentiment d'inquiétude résultant de l'orientation prise par la construction intercommunale depuis les lois Maptam et NOTRe. Sur le terrain, de plus en plus de voix s'élèvent en effet pour nous dire que l'esprit n'y est plus, ce que vous avez d'ailleurs rappelé, monsieur le ministre. Les élus municipaux ont le sentiment d'être pris dans de vastes ensembles, et parfois décrochent. Sans surprise, la question de la gouvernance des EPCI revient comme un serpent de mer. Les élus municipaux communautaires et,, les élus non communautaires, estiment qu'ils ne sont pas toujours suffisamment ou correctement bien associés aux décisions de l'intercommunalité. Cette réalité a été confirmée par les résultats de la consultation que nous avons lancée le 27 mars dernier sur la place des élus municipaux dans la gouvernance des intercommunalités, que certains d'entre vous ont bien voulu relayer auprès des élus dans les territoires. Soyez-en remerciés, car nous avons déjà obtenu plus de 4 000 réponses en seulement trois semaines d'enquête. Cela témoigne de l'intérêt du sujet pour les élus municipaux

Les règles de représentation au sein des conseils communautaires sont elles aussi souvent critiquées. Dans cette perspective, la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui va dans le bon sens. Le bon fonctionnement des EPCI nécessite effectivement une parfaite coordination entre les conseils municipaux et les conseils communautaires. Comme le relève opportunément le rapporteur de la commission des lois, il s'agit, d'une part, d'une « condition de la légitimité de l'action communautaire » et, d'autre part, d'« un gage de bonne administration locale tant les compétences communales et intercommunales sont étroitement imbriquées. Je suis surtout heureux que ce texte, modifié par la commission des lois, tende à mieux associer les maires au fonctionnement quotidien des EPCI, notamment grâce à l'instrument de la conférence des maires.

mettre fin au suspense, les deux grands objectifs de ces recommandations destinées à faire place aux bonnes pratiques de gouvernance au sein des instances communautaires il s'agit, d'une part, de mieux associer l'ensemble des conseillers communautaires aux décisions de l'EPCI et, d'autre part, d'associer plus systématiquement les élus municipaux non communautaires à ces décisions. Vous l'aurez compris, notre but est de favoriser l'implication des élus municipaux dans le fonctionnement des intercommunalités. sein de la délégation aux collectivités territoriales, sous l'égide de notre président Jean-Marie Bockel, nous avons choisi une approche originale et consensuelle : nous avons identifié les outils déployés dans les territoires pour répondre à cet objectif d'associer pleinement les élus municipaux à la vie et à la gouvernance des EPCI. Notre travail a donc essentiellement visé à valoriser ces bonnes pratiques qui méritent d'être diffusées. C'était d'ailleurs une revendication très forte des acteurs de terrain que nous avons auditionnés et que nous avons rencontrés lors de nos déplacements faire confiance à l'intelligence territoriale, faire preuve de souplesse et n'imposer aucun carcan législatif, tels sont les messages qu'ils nous ont adressés. Comme l'affirmait le président du Sénat en novembre dernier lors du colloque de la commission des lois, consacré au rapport de notre collègue Mathieu Darnaud visant à revitaliser l'échelon communal, tout n'est pas du domaine législatif » et « c'est le rôle du Sénat que de mettre en lumière les bonnes pratiques ». À la délégation aux collectivités territoriales, nous nous sommes inscrits dans cette démarche- n'est-ce pas, chère Françoise Gatel ? En effet, il n'existe pas de solution unique. Les réponses, les outils, les pratiques peuvent varier d'un territoire à un autre, d'un EPCI à un autre. Reste l'objectif fondamental : replacer l'élu municipal au coeur de la démocratie intercommunale. Je me félicite de ce que, dans les différentes instances du Sénat, et quelles que soient nos sensibilités politiques, les avis convergent pour faire en sorte

centaine d'heures de débats avec le Président de la République, et surtout qui ai les pieds dans la glaise de mon département de coeur et d'élection, l'Eure, je dois avouer que je ne sais pas très bien quelle question supplémentaire il faut poser aux élus locaux sur leur appréciation de la loi NOTRe. En revanche, vous avez raison

pas diagnostiqués. Comme je vous l'avais dit lors de la discussion du projet de loi de finances, il nous faut rouvrir cette question globale de l'organisation territoriale en Île-de-France et au sein de la métropole du Grand Paris.

mais également pour les entreprises et celles et ceux qui investissent sur le territoire du Grand Paris. C'est un chantier que nous aurons à connaître dans les semaines et les mois prochains. Du retard a été pris, je ne dis pas le contraire, mais une fois de plus, si c'était simple, ça se saurait

toutes les ressources au détriment du monde rural. Mais il ne faut pas non plus des intercommunalités de 5 000 habitants dans le monde rural qui n'ont pas l'efficacité nécessaire. De nombreux élus se sont dotés d'intercommunalités, de communautés de communes ayant une certaine taille critique, donc pouvant se doter, monsieur le ministre,

qu'il ne faut pas être forcément adjoint pour être délégué à l'intercommunalité. Très franchement, je ne vois pas pourquoi on a retenu ce mode de désignation parfaitement tordu,

Il concerne une défaillance temporaire du maire : si un maire ne peut pas se rendre temporairement à un conseil communautaire, son suppléant

en rétablissant le principe selon lequel les conseils municipaux élisent leurs délégués en leur sein, mais cette fois, dans les seules communes de moins de 1 000 habitants. Comme vous le savez, les conseillers communautaires de ces petites communes sont désormais dans l'ordre du tableau du conseil municipal. Cette règle a été adoptée par analogie avec le système du fléchage dans les communes de plus de 1 000 habitants, puisque, en dehors du maire et des adjoints, le rang des simples conseillers municipaux dans l'ordre du tableau dépend du nombre de suffrages qu'ils ont obtenus lors des élections. Un lien est ainsi établi avec le suffrage universel. Il ne me semble pas opportun de revenir en arrière, au risque de fragiliser l'équilibre trouvé en 2013.

l'ordre du tableau, tout en permettant l'exception, la souplesse que j'indiquais tout à l'heure lors de ma très longue intervention. D'ailleurs, j'ai fait fuir le ministre Sueur, ce qui est bien dommage. Le Sénat reproche au Gouvernement de ne pas être suffisamment disponible pour lui, mais, quand je me montre disponible

pourquoi ne pas revenir à la méthode la plus simple, la plus claire : le conseil municipal désigne à la fois les adjoints et les délégués

reposer les décisions qui ont été prises antérieurement, car les équipes municipales se sont familiarisées avec ce mode de désignation. Nous savons tous que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, la présentation de la liste prendra en considération les modes de désignation à l'intercommunalité, et ce sans aucun problème. Il faut donc laisser un peu de temps au temps.

de l'impossible. Il s'agit non pas de laisser reposer en paix de manière définitive les irritants de la loi NOTRe, mais de trouver des solutions en gardant une cohérence et une sorte de colonne vertébrale.

Dans les communes ne disposant que d'un siège au conseil communautaire, un conseiller suppléant est désigné, ce qui permet à la commune d'être représentée en l'absence ponctuelle du conseiller élu, qui est généralement le maire. le maire. M. Gremillet propose que, en cas d'empêchements simultanés du conseiller titulaire et du conseiller suppléant, un autre membre du conseil municipal puisse être appelé à siéger à leur place, selon des modalités définies par décret. Je comprends bien qu'il s'agit de remédier à des problèmes pratiques qui se posent sur le terrain. Néanmoins, ces dispositions soulèvent deux difficultés. Premièrement, le législateur ne peut pas renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir les règles de suppléance dans les assemblées locales : c'est le coeur du fonctionnement démocratique des assemblées locales qui est en jeu,

métropolitains au suffrage universel. À ce titre, le Gouvernement devait présenter un texte de loi avant le 1 janvier 2019 : il ne l'a pas fait, sans pour autant

est à M. Stéphane Artano. La conférence des maires, prévue au présent article, est inspirée de la proposition n° 23 du rapport d'information sur la revitalisation de l'échelon communal du 7 novembre 2018, visant à mieux associer les maires au fonctionnement de l'intercommunalité.

De même, la commission a prévu que la demande de création d'une conférence des maires devrait être formulée dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Il ne me paraît pas souhaitable de supprimer cette condition : le système de gouvernance fixé doit être défini pour toute la durée de la mandature.

la représentation démocratique et, partant, démographique. Le conseil communautaire tient compte du poids de la population : c'est un principe de base qu'il est important de rappeler.

part d'une bonne intention. À titre personnel, je souhaite d'ailleurs que les conférences des maires deviennent obligatoires. Certes, plus de 70

La conférence métropolitaine est une instance consultative qui regroupe tous les maires de la métropole ; en 2020, il s'agira du seul organe où les communes seront représentées.

« conférence métropolitaine des communes », afin de souligner le fait que les communes sont associées pleinement à la gouvernance de la métropole de Lyon.

ou le schéma métropolitain des solidarités. Quel est l'avis de la commission ? La commission a prévu que les projets d'actes les plus importants de la métropole et ceux qui se rapportent le plus étroitement aux compétences communales

Nos collègues proposent d'y ajouter les projets de schéma métropolitain des solidarités, de schéma métropolitain éducatif et culturel ainsi que le projet de programme métropolitain d'insertion par l'emploi.

En outre, pour contourner ses obligations de consultation, il suffirait à la métropole de cesser d'élaborer ces schémas et ces programmes. Avis défavorable.

de grandes communes de la métropole de Lyon, pourraient ne pas siéger au conseil métropolitain, alors même que leurs opposants,

se donnerait l'objectif de contrecarrer les effets de la création de la métropole en tant que collectivité locale élue au suffrage universel direct

des communes membres d'un même bassin de vie. Dans le pacte métropolitain, elles sont présentées comme des instances de concertation. Pour autant, aujourd'hui, elles ne fonctionnent pas,

Elles auront ainsi l'occasion de débattre de l'exécution des politiques métropolitaines à l'échelle des bassins de vie et deviendront des lieux d'échanges et de discussions pour permettre une bonne adaptation des politiques métropolitaines au niveau communal. Quel est l'avis de la

Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques de la métropole. Nos collègues proposent que leur consultation soit désormais obligatoire. J'y suis très J'y suis très défavorable, pour des raisons de droit et d'opportunité. Tout d'abord, cet amendement, tel qu'il est rédigé, tend à exiger que chacune des conférences territoriales des maires soit consultée, à peine de nullité, sur chacun des projets d'actes de la métropole, ce qui risquerait de paralyser son fonctionnement et de provoquer des annulations en série, dans le cas où cette formalité ne serait pas systématiquement accomplie. ces conférences territoriales ne doivent pas nécessairement être toutes consultées sur tous les sujets, mais seulement sur les politiques métropolitaines qui concernent spécifiquement leur territoire. Pour que les communes soient associées à l'élaboration des politiques conduites sur l'ensemble du territoire métropolitain, il existe une autre instance : la conférence métropolitaine. Il ne me paraît pas non plus indispensable de fixer, pour ces conférences territoriales, un minimum d'une réunion par semestre au lieu d'une réunion par an. Les élus ont parfois autre chose à faire que de multiplier les réunions. En cas de nécessité, une réunion peut toujours être convoquée sur l'initiative du président de la conférence territoriale, qui est un maire, ou de la moitié de ses membres. Avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement

des funérailles républicaines, un débat sur ces deux valeurs : liberté d'un côté, égalité de l'autre. J'entends que vous êtes soucieux qu'une égalité soit constatée sur la manière dont sont organisées la vie locale et la démocratie au sein de la métropole de Lyon.

la métropole de Lyon, des questions institutionnelles sont « encore en suspens ». En 2014, l'élection des conseillers communautaires concernait 59 communes

Ainsi, il est prévu que les 166 " conseillers métropolitains de Lyon sont élus dans chacune des circonscriptions métropolitaines au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. " » Ils ont rencontré les élus, y compris les maires, Dans la mesure où, d'une part, il n'y aura plus de fléchage, mais un scrutin par liste et où, d'autre part, dans certaines circonscriptions, le nombre d'élus est inférieur au nombre de communes, certaines d'entre elles ne seront plus représentées au sein du conseil métropolitain. » Ils citent ensuite l'exemple de la circonscription métropolitaine Val-de-Saône à laquelle sont attribués

Comme vient de le rappeler ma collègue Annie Guillemot, nous représentons à la fois le « nouveau Rhône » et la métropole de Lyon et nous avons des relations avec les maires des municipalités qui constituent

ceux qui ont assisté au débat sur la création de cette merveilleuse institution qu'est la métropole de Lyon se rappellent quelles étaient les bonnes fées autour du berceau.

Je suis un peu dubitatif quant à l'intérêt de cette mesure. Les grandes lignes du projet politique des candidats auront été exposées durant la campagne électorale ; pour le reste, le président de l'EPCI ne dispose pas toujours de la visibilité nécessaire pour élaborer un programme détaillé des actions à mener

ne prend pas la parole dans la presse pour expliquer ce qu'il veut faire au sujet des compétences qu'il a acquises de par la loi ou la volonté locale, s'il n'informe pas les maires, les conseillers communautaires et les conseillers municipaux de sa vision politique,

avec un document un peu scolaire ou un rapport que l'on enverrait à tous les conseillers municipaux pour expliquer ce que l'on va faire ? Cela s'appelle une profession de foi électorale et, une fois de plus, un EPCI n'est pas une collectivité territoriale- je mets le cas de Lyon de côté. de côté. Où faut-il s'arrêter ? Madame Lherbier, enfin, ce que vous proposez s'appliquera autant à une communauté de communes rurales du département du Nord qu'à la métropole de Lille. Reconnaissez que la vie démocratique n'y est pourtant pas forcément organisée de la même manière ! Très bien

est à M. François Bonhomme.

lundi 15 avril, quelques heures seulement après le déclenchement du grand incendie de Notre-Dame, la communauté internationale se mobilisait déjà pour soutenir la reconstruction de la cathédrale. En quelques jours, près de 1 milliard d'euros de dons ont été collectés, un projet de loi annoncé et un vaste plan de reconstruction mis en ordre de bataille. Loin devant la collecte du loto du patrimoine, cet élan de générosité intervient après un certain nombre d'années de forte baisse des ressources publiques consacrées au patrimoine, dont l'entretien et la restauration reposent en grande partie sur les communes. À l'heure de la programmation de ce débat au Sénat, nous ne savions pas que l'actualité allait mettre de cette façon le mécénat territorial sous les feux de la rampe. Nous voulions avant tout susciter une réflexion de fond sur le développement du mécénat en faveur de nos collectivités Celles-ci sont de plus en plus nombreuses à lever des fonds auprès d'acteurs privés pour financer des projets locaux. Selon l'étude menée conjointement par Ernst&Young et Régions de France, si les sommes en jeux restent modestes, le potentiel de développement est bien réel. Ainsi, la Folle journée de Nantes, terrain d'innovation artistique et culturelle, est soutenue par un réseau de mécènes qui ont permis de lever 2,8 millions d'euros en 2015. Dans le même esprit, la région Nouvelle-Aquitaine a mis en service une plateforme de financement participatif sur laquelle il est possible de soutenir des projets variés, du financement d'ateliers intergénérationnels au développement d'une marque d'artisans et de producteurs régionaux. Alors que les collectivités territoriales n'hésitent plus à lancer des campagnes de souscription pour acquérir une oeuvre, rénover un monument ou contribuer au financement des initiatives citoyennes, il serait dommage de voir dans le mécénat territorial un simple moyen de compenser la baisse des concours de l'État, évaluée à 9,6 milliards d'euros depuis 2014. L'État n'a pas le monopole de l'intérêt général. dite loi Aillagon, a opéré un changement de dialectique entre solidarité nationale et mécénat, offrant une vraie reconnaissance à l'ensemble des acteurs mobilisés en faveur de l'intérêt général. La loi de 2007 étend cette reconnaissance aux monuments historiques privés, aux organismes du spectacle vivant et ouvre une dimension européenne aux actions de mécénat. La France s'est ainsi dotée d'un dispositif fiscal parmi les plus avantageux au monde en faveur du mécénat. En 2017, le mécénat d'entreprise représentait en France 3,5 milliards d'euros de dons. Le nombre d'entreprises mécènes et de fondations progresse année après année. Reste que ce qui est une évidence dans la culture anglo-saxonne l'est beaucoup moins en France, où la philanthropie a longtemps été éclipsée par la sphère publique. Tandis que l'espace démocratique semble parfois se réduire aux élections, qui restent les grands jalons de la vie démocratique, les mouvements sociaux que nous traversons témoignent d'un besoin d'horizontalité, de proximité, de participation plus directe aux projets locaux, permettant à chaque citoyen de trouver sa place au sein de la collectivité. Le dispositif actuel n'est pas sans faille. En 2016, 24 entreprises ont réalisé 44 % de la dépense fiscale au titre de la loi sur le mécénat. Les phénomènes de concentration, en termes tant d'entreprises bénéficiaires que de répartition territoriale des projets, posent un certain nombre de questions. finances, d'un plafond en valeur des dons ouvrant droit à réduction d'impôt contribuera, nous l'espérons, à favoriser le développement du mécénat des petites entreprises. Les collectivités territoriales n'en sont pas les premières bénéficiaires, bien que de plus en plus d'entreprises soutiennent des structures publiques. Nous pensons que le développement du mécénat territorial est une chance pour la France. En fédérant un réseau de mécènes autour de projets locaux, ce levier de développement est à la fois un vecteur d'identité et de cohésion territoriale, un moyen de communication complémentaire, offrant de la visibilité aux projets, et une façon de retrouver un certain élan démocratique à travers une participation directe et concrète des citoyens et des entreprises. Alors que cette nouvelle voie doit encore monter en puissance, le débat de cet après-midi nous permettra d'échanger autant sur les opportunités d'une telle démarche pour les collectivités que sur les obstacles qu'elles rencontrent encore pour développer leurs propres initiatives de mécénat. Au premier rang de ces obstacles figurent le manque de professionnalisation, donc d'expertise, des collectivités territoriales en la matière, l'insécurité juridique qui résulte des changements ou perspectives de changements trop fréquents dans la réglementation et la méconnaissance, voire l'ignorance du dispositif par les collectivités territoriales elles-mêmes. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le mécénat territorial est une forme de réponse l'expression de forces centrifuges de dissolution du lien local : fusion des régions, montée en puissance des intercommunalités, concentration des pouvoirs et éloignement des centres de décision. Les liens qui hier encore nous rassemblaient se distendent aujourd'hui. Il nous appartient de redonner du sens à l'action locale et de permettre à chacun de trouver sa place dans une société trop diluée, confuse, défiante, à travers ce facteur de concorde que représentent le mécénat

Ce sujet est particulièrement sensible dans le contexte actuel de la rénovation de Notre-Dame de Paris, qui ne saurait toutefois résumer à elle seule l'action de l'État et des collectivités territoriales J'ai accompagné le Président de la République dans sa grande consultation des maires : j'ai pu constater, une fois de plus, à quel point les questions de proximité et d'enracinement sont au coeur des préoccupations des citoyens et des élus locaux,

Au fond, qu'est-ce que le mécénat territorial, notion qui n'a pas de définition juridique ? Il s'agit d'un dispositif fondamentalement interministériel, piloté au ministère de la culture, mais aussi au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et surtout à Bercy, compte tenu des montants en jeu- j'y reviendrai. Le mécénat territorial revêt, avant tout, une dimension de compétences : il s'agit de savoir comment mobiliser des ressources humaines d'entreprises, de particuliers ou d'autres collectivités au service de projets d'intérêt général. Ensuite, le mécénat territorial revêt une dimension financière : comment réussir à lever des fonds privés et à les associer à des fonds publics au service de projets d'intérêt général sur les territoires ? Qu'est-ce qui explique le recours au mécénat territorial ? Premier constat : il a été encouragé ces dernières années par l'ampleur du chantier de rénovation à conduire. la France compte des centaines de milliers de bâtiments dignes d'intérêt. La rénovation de ces bâtiments est cyclique, et les besoins ne cessent de s'accroître. Les ministères sont de longue date impliqués aux côtés des collectivités propriétaires de la moitié des 44 000 immeubles historiques protégés, dans l'effort de rénovation du patrimoine. Deuxième constat : la baisse de la DGF entre 2013 et 2017 a encouragé le recours au mécénat territorial.

La mobilisation de plus de 300 millions d'euros chaque année par ce ministère en faveur de la conservation des monuments historiques correspond à une augmentation de 5 %. Le loto du patrimoine, piloté par Stéphane Bern, a été un succès, avec 20 à 25 millions d'euros de fonds récoltés supplémentaires. Il s'ajoute à de nombreuses initiatives innovantes, comme le financement participatif. En 2018, le comité de sélection a retenu 269 édifices appartenant surtout à des propriétaires publics. La répartition géographique des projets sur l'ensemble du territoire a été prise

est ainsi le plus avantageux d'Europe. L'élan de générosité des entreprises comme des particuliers auquel on assiste depuis l'incendie qui a gravement endommagé la cathédrale Notre-Dame de Paris en est une des manifestations les plus éclatantes. À un événement d'exception, nous avons répondu par un dispositif d'exception. En 2017, quelque 3,8 milliards d'euros

Le montant des dons a augmenté de 380 % depuis 2004 : il représentait alors 1 milliard d'euros. Ce mouvement devrait se poursuivre avec la modification du plafond de défiscalisation dans la loi de finances de

a été remis en novembre dernier. Des réflexions sont en cours sur ces dispositifs, sur la base de ce rapport. Toutefois, la position du Gouvernement est de veiller à ne pas introduire de modifications fiscales majeures dans un dispositif qui a fait ses preuves et qui continuera à faire ses preuves. Enfin, des réflexions sont engagées pour favoriser le mécénat de compétences, car de trop nombreux freins existent encore. Même si celui-ci est encadré par le droit européen de la concurrence, nous pouvons probablement apporter plus de souplesse au cadre existant. Nous pouvons, par exemple, aller plus loin en permettant plus facilement à un citoyen bénévole de s'investir dans un projet d'intérêt général, à l'image des journées citoyennes organisées dans un certain nombre de territoires. Nous pouvons aussi aller plus loin dans l'assistance technique ou l'exercice en commun de compétences entre les collectivités. Sur ce point, je communiquerai d'ici à la fin du mois un guide des mutualisations. Nous pouvons enfin aller plus loin en favorisant le mécénat de compétences de la part d'entreprises privées. Il n'y en a pas assez ! Des discussions sont d'ailleurs en cours dans le cadre de la proposition de loi sur l'Agence nationale de la cohésion des territoires, portée par Jacqueline Gourault. rapidement plus de souplesse au cadre existant. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que je souhaitais vous indiquer en introduction de nos débats sur cet important sujet, qui doit tous nous mobiliser.

Or ce patrimoine, témoin de l'histoire de nos régions, de notre histoire, est en danger. Depuis plusieurs années, nos collectivités locales débordent d'imagination pour favoriser le mécénat territorial, avec succès. Des partenariats entre entreprises mécènes et collectivités ont ainsi émergé et permis de réaliser de grandes avancées en matière de sauvegarde du patrimoine local. Le véhicule juridique privilégié par les collectivités est généralement le fonds de dotation. Or ce dernier présente actuellement une limite majeure puisque la collectivité a interdiction de l'abonder. Cette mesure contraint le fonds de dotation à affecter une part de la collecte au financement des dépenses de fonctionnement. Cette situation est pénalisante dans un contexte d'émergence de cette forme de mécénat, car les montants de collecte sont parfois encore modestes. Autoriser les collectivités à abonder ce fonds lui permettrait de se constituer une dotation d'amorçage et d'absorber une part des coûts de fonctionnement par la mise à disposition de personnels ou de locaux. Monsieur le ministre, comptez-vous légiférer sur ce point, afin de permettre aux collectivités territoriales d'abonder les fonds de dotation en vue de favoriser le mécénat et ainsi la sauvegarde du patrimoine local ? La parole est à M. le ministre.

à la main du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics pour des situations particulières, sans qu'il soit, à mon avis, besoin de modifier le cadre législatif global. Voilà ce que je puis vous dire en moins d'une minute.

Mais, voyez-vous, la fin de la réserve parlementaire a dû nous rendre plus créatifs pour ce qui concerne le soutien du patrimoine local. Le département de l'Orne a mis en place, un peu sur mon initiative, un fonds de dotation pour le patrimoine.

ne peut pas servir à nourrir les opérations que nous voudrions soutenir.

Je l'ai vu dans un département voisin, l'Eure, l'expertise d'ingénierie en bâtiment est un énorme enjeu. Certes, les services du ministère de la culture sont là

parfois un peu risqué sur le plan juridique. Voilà encore une piste intéressante : une mairie importante a des ingénieurs en bâtiment ; une commune rurale a un projet pendant le mandat de son maire ou pendant dix ans. Comment le maire de la commune-centre, le président de la communauté d'agglomération ou le président du conseil départemental

monsieur le ministre, mes chers collègues, je vis dans un département qui compte plus de 1 000 églises. C'est non seulement une richesse, mais également une lourde charge pour les petites communes qui en sont propriétaires et, à ce titre, en assument l'entretien et la préservation. À ces églises s'ajoute souvent un petit patrimoine dit « vernaculaire Ces deux patrimoines, les églises et le « vernaculaire », peinent à trouver leur place face à notre « glorieux » patrimoine. Ils sont souvent mal protégés et peuvent se retrouver parfois à l'abandon. Une réhabilitation est difficile et coûteuse. coûteuse. Les petites communes rurales n'ont que des priorités, compte tenu de la modestie de leur budget : l'école, la mairie, la voirie, le cimetière, l'éclairage public, et j'en oublie certainement. Dans nos territoires ruraux, ces patrimoines riches et anciens présentent pourtant de nombreux avantages. C'est l'identité des villages et de la ruralité qui est en cause : l'église, le monument aux morts, le lavoir, le puits, le moulin, la mare sont les reliques d'un passé qui a du sens, et ils caractérisent l'authenticité de la ruralité. Entretenir ce patrimoine, c'est assurer bon an mal an des travaux de maçonnerie, de peinture, de menuiserie, de couverture. Cela fait donc vivre l'artisanat local ; ce n'est pas rien ! Enfin, ces patrimoines présentent une richesse touristique qui, restaurée et mise en valeur,

Particuliers et entreprises ont un rôle déterminant à jouer, vous l'avez dit, pour valoriser nos richesses. Dans mon département du Nord, à Tourcoing- vous le savez, j'aime en parler -, le musée des Beaux-Arts a pu bénéficier d'un partenariat solide des entreprises locales le mécénat. Une grande exposition sur les chrétiens d'Orient a pu voir le jour et a eu un immense succès grâce à ces entreprises locales. C'est une façon de communiquer pour elles du « gagnant-gagnant » pour nos territoires et nos acteurs économiques, qui jouissent dès lors tous deux d'une bonne image. Mais la portée du mécénat ne s'arrête pas à la protection du patrimoine ou à la promotion culturelle. C'est aussi un moyen efficace pour mener des actions sociales. Toujours à Tourcoing, l'action « 1 livre, 1 enfant » permet, grâce au mécénat, la distribution de livres à tous les enfants des écoles, favorisant ainsi le développement culturel, notamment dans les quartiers difficiles. Ces actions sociales sont souvent vitales pour revitaliser les zones rurales et aider les populations qui se sentent abandonnées par les pouvoirs publics. Comment comptez-vous soutenir ces initiatives et faire en sorte que cette dynamique se perpétue ? dynamique se perpétue

de confier de l'argent à une collectivité territoriale pour une opération de rénovation, pour un projet culturel, il entend que l'environnement normatif, législatif, réglementaire

ainsi. Il s'agit pour elles de participer ainsi aux infrastructures publiques. Mais, ne soyons pas naïfs ! La réduction substantielle d'impôt et la possibilité de choisir

citoyenne dans le fait de participer à un projet. Les entreprises concernées ne sont pas que les grandes entreprises ; il y a aussi des entreprises de proximité. On a beaucoup parlé de culture et de patrimoine depuis tout à l'heure, mais le sport entre également dans le champ du mécénat territorial.

Monsieur le président, messieurs les ministres, le mécénat permet entre autres l'aboutissement de projets en lien avec les territoires. En cette période où les ressources financières des collectivités sont fragilisées, cette voie est donc à privilégier. Dernièrement, nous avons vu avec peine un chef-d'oeuvre architectural, un symbole fort de notre histoire, en proie aux flammes. Mais, malheureusement, combien de monuments, combien de sites historiques et culturels, chargés de valeur, sont au bord de l'effondrement ? Combien de patrimoines à préserver davantage sont à dénombrer dans nos nombreuses communes ? Les exemples se multiplient tristement. Aussi, la France dispose d'un cadre fiscal assez attractif, qui permet de favoriser ce mode de financement. Cependant, parmi les difficultés qui existent, il y a celle de la mise à disposition, et plus généralement celle du manque d'information sur les manières de contribuer. Dans plusieurs cas, nous avons observé l'existence de plusieurs plateformes consacrées à la collecte de fonds. Je veux croire qu'elles partent d'un bon sentiment. Toutefois, des citoyens, mais aussi des acteurs privés ou publics pourraient parfois être victimes d'une forme de confusion face à la multiplication de ces supports, comme les cagnottes en ligne, en particulier lorsqu'un traitement médiatique d'envergure nationale a été consacré à un bien connu. Cette confusion est d'autant plus importante quand nous apprenons l'existence de manoeuvres frauduleuses, ce qui renforce alors le sentiment d'insécurité. Ainsi, ne serait-il pas envisageable, monsieur le ministre, de créer, par exemple, une plateforme unique officielle, qui aurait pour objet de répertorier chaque support créé pour participer à des projets nationaux et locaux Une telle possibilité faciliterait la mise à disposition, sur un site public et sécurisé, d'informations vérifiées. Nous pourrions également imaginer un système où les dons publics seraient indiqués. En outre, un tel site favoriserait la transparence et la traçabilité des donations publiques. Bien évidemment, je parle de « mise à disposition » ; il ne devrait en aucun cas s'agir d'une mainmise de la puissance étatique sur le mécénat ni d'un contrôle. Par conséquent, est-il possible, monsieur le ministre, de recueillir l'avis du Gouvernement sur cette proposition et de connaître plus généralement les pistes envisagées pour pallier les difficultés que je viens de soulever ? La parole est à M. le ministre. Monsieur le

On peut se réjouir de ce vote en ce 9 mai, qui célèbre la Journée de l'Europe. C'est une belle satisfaction que de voir que la France est le premier pays à avoir transposé la directive sur le droit d'auteur pour laquelle elle s'est beaucoup mobilisée avec les parlementaires européens.

1 000 euros, sachant que les règles s'appliquant aux entreprises pour le mécénat restent inchangées. À cet égard, nous avons voulu rassembler les trois fondations et l'institution dans un même portail pour garantir

de la culture, qui nous a rejoints. Il y a trois ans, lors de l'examen du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la loi LCAP, le Sénat avait proposé une nouvelle forme de mécénat territorial. Le rapporteur du texte pour la commission de la culture, M. Jean-Pierre Leleux, avait alors suggéré de mettre en place un dispositif permettant aux entreprises et aux commerçants d'une commune ou d'une intercommunalité de soutenir l'action d'un organisme associatif

On pourrait prévoir que la déduction fiscale sur la cotisation foncière des entreprises, impôt local payé soit à la commune, soit à l'EPCI, soit limitée à 60 %, comme dans les dispositifs nationaux, et plafonnée, par exemple à 2 500 euros par don. Il n'y aurait bien évidemment aucune obligation pour les collectivités à mettre en oeuvre le dispositif proposé. Je crois beaucoup à une implication territoriale du mécénat, à la proximité. Les collectivités connaissent, nous le savons, les entreprises de leur territoire. Dans un contexte de baisse des dotations, comme cela a été rappelé, cela leur donnerait la possibilité d'optimiser des ressources extérieures. Nous avions adopté ce dispositif lors de la discussion de la loi LCAP, mais la ministre Fleur Pellerin, bien que favorable sur le principe, souhaitait qu'une expertise soit menée. Monsieur le ministre, cette expertise a-t-elle bien eu lieu ? Que pensez-vous de cette proposition ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai la chance de représenter au Sénat un département, le Calvados, qui est l'un des plus riches de France en matière patrimoniale. Il se classe même au troisième rang national pour ce qui est du nombre des monuments historiques, inscrits ou classés, qui embellissent villes et campagnes d'une architecture variée et participent à l'attractivité touristique. Tout le monde sait que, depuis la loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État, l'entretien des églises et chapelles construites avant cette date ainsi que celui des oeuvres communes qui en sont propriétaires. À l'heure où les mécènes se sont rapidement mobilisés pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, il me semble opportun d'évoquer l'entretien du patrimoine religieux de nos petites communes rurales. Bien sûr, il y a les dons des fidèles, mais ce n'est pas suffisant. On me dira qu'il existe des dotations du ministère de la culture, qu'un fonds incitatif et partenarial pour les monuments historiques situés dans les communes à faibles ressources a été reconduit en 2019 ou que les départements et régions peuvent également intervenir. De toute évidence, je le répète, cela ne suffit pas pour faire face aux besoins actuels. La mise en place de démarches structurées de mécénat fait encore figure d'innovation au sein de nombre de collectivités, en particulier en milieu rural. nécessitent une adaptation tant des élus et des agents que des parties prenantes externes, les TPE-PME n'étant pas toujours au fait des incitations prévues par la loi Aillagon de 2003. Il convient donc d'encourager une forme de professionnalisation des différents acteurs et l'échange de bonnes pratiques.

Les collectivités territoriales sont aussi légitimes que n'importe quelle structure pour porter des projets de mécénat. Je rappelle que 81 % des entreprises disent privilégier des projets au niveau local et régional et 71 % des fondations et fonds de dotation tiennent compte des lieux d'implantation géographique de leur entreprise au moment de la sélection des projets. Autre chiffre intéressant, environ 85 % des entreprises ne font pas appel au mécénat. Cela laisse donc d'immenses possibilités de développement. Encore faudrait-il que le dispositif soit clair et encourage les acteurs locaux à s'engager dans cette démarche sur leur territoire

Dans le même sens, en juillet 2018, la mission d'information sur le mécénat culturel conduite par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat en appelait, dans ses conclusions, au développement du mécénat territorial. Selon les conclusions de cette mission d'information, les entreprises seraient désormais « plus plus mûres pour cette évolution, compte tenu de leur attrait pour des projets de proximité ». Qu'en est-il de la mise en application ? À l'occasion de leurs travaux, nos collègues ont notamment pu relever que, si les DRAC

leurs correspondants mécénat font parfois face à des manques de moyens ou de personnels évidents. Dans certaines situations, les DRAC se contentent d'un rôle plutôt technique, qui porte notamment sur les autorisations de travaux et les études préliminaires. La gestion du mécénat revient alors aux collectivités et nombreux sont les départements qui sont appelés à s'organiser avec les moyens du bord ... Dans leurs conclusions, nos collègues de la mission d'information sur le mécénat culturel invitaient à ce titre l'ensemble des collectivités à se saisir de cette problématique afin d'éviter que les inégalités ne se creusent davantage.

pour écrire les statuts, prospecter et convaincre les entreprises de s'inscrire dans le projet. Par ailleurs, au-delà de la collecte des dons, il faut trouver des porteurs de projets suffisamment organisés et solides, capables de mettre en oeuvre des initiatives susceptibles d'attirer les capitaux privés.

le ministre, nos territoires ont besoin d'un tissu associatif dynamique qui permet, au travers de l'activité des bénévoles, de créer et d'entretenir le lien social. Le sport, dont nous avons peu parlé jusqu'à présent, est une activité déterminante de ce point de vue. Le développement d'activités physiques et sportives pour tous souffre de problèmes financiers non négligeables, mais également de difficultés en termes de ressources humaines. Un soutien plus important, à l'échelon local, du monde de l'entreprise, de l'artisanat et du commerce est souvent demandé par les associations, notamment au travers du mécénat. Dans les territoires, ce dispositif est souvent confondu avec le sponsoring. Il est donc nécessaire de mieux faire connaître ces dispositifs et de les sécuriser pour éviter tout redressement fiscal.

les échanges qui ont nourri notre débat ont démontré que le mécénat territorial au service des projets de proximité est amené à se développer. Ils ont également confirmé le fait que les collectivités territoriales sont encore loin de s'être approprié ce dispositif. Un soutien public à l'initiative privée, voilà ce qu'est le mécénat. Mieux, je crois que le dispositif constitue également un outil de cohésion territoriale. Le groupe Les Indépendants a déposé une proposition de loi en ce sens. Elle vise à engager plusieurs actions au niveau national pour diffuser plus largement les pratiques du mécénat auprès des collectivités territoriales. Mais l'action ne doit pas seulement viser les collectivités. La France a besoin d'entrepreneurs mécènes, qui ne se contentent plus de leur rôle économique, mais orientent leurs actions vers des projets à vocation sociale, environnementale, culturelle ou sportive. C'est le sens de la journée nationale de la philanthropie que nous appelons de nos voeux sur le modèle de ce qui se pratique chaque année aux États-Unis. C'est également le sens du label Entreprises engagées, que nous voudrions attribuer à toutes les entreprises qui donnent un montant égal à cinq pour mille de leur chiffre d'affaires Le groupe Les Indépendants souhaite porter l'ambition d'inventer une nouvelle philanthropie à la française. Il s'agit de reconstruire la relation des citoyens à la chose publique, en leur permettant d'orienter la dépense publique vers les projets qu'ils considèrent comme prioritaires au niveau local. Nous en